Cet amendement n'est pas que symbolique, dans une période où le pouvoir d'achat est l'une des problématiques prioritaires de nos concitoyens. Il vise à exonérer toutes les pensions de retraite et d'invalidité, et pas seulement les plus modestes, de l'augmentation de 1,7 point du taux de la CSG applicable depuis le 1janvier 2018. Depuis cette date, les retraités ont subi cette hausse, mais ils s'apprêtent aussi à subir en 2019 une sous-indexation de leurs pensions. Comme on dit trivialement : ils l'ont senti passer ! Ils nous l'ont dit sur le terrain, et ils le disent aux ministres ou au Président de la République, quand ils ont l'occasion de le croiser. Eux qui ont travaillé, cotisé toute leur vie, eux qui incarnent la solidarité intergénérationnelle, en aidant leurs enfants, leurs petits-enfants et leurs parents dépendants,

morale. La relance de l'économie grâce au travail est une évidence- c'est le discours du Président de la République -, mais elle ne doit en aucun cas être menée au détriment de ceux qui ont façonné le monde d'aujourd'hui par leur travail d'hier, et qui ont encore beaucoup à apporter.

L'augmentation de la CSG de 1,7 point sur les retraites et sur les pensions d'invalidité va évidemment porter atteinte au pouvoir d'achat de 7,5 millions de retraités. Cette hausse de la CSG correspond en fait à une augmentation de 25 % pour 9 millions de retraités, soit une ponction directement dans leurs porte-monnaie de 4,5 milliards d'euros par l'État. Seuls les retraités percevant plus de 1 200 euros net par mois sont théoriquement concernés par cet effort en faveur des salariés. Or il faut savoir que le plafond en dessous duquel les retraités échappent à la hausse de la CSG est basé non pas sur la retraite, mais sur le revenu fiscal de référence 2016, dont le montant pour 2018 a été arrêté à 14 404 euros pour une part de quotient familial, soit 1 200 euros net par mois, ce qui veut dire que ce barème peut très vite être dépassé selon la situation familiale. quelques exemples donnés par le journal, dans son édition du 21 septembre dernier. Anne, ancienne infirmière, perçoit 970 euros net de retraite et son mari Jean, ancien employé municipal, 1 010 euros net. Tous deux, en limite du seuil de pauvreté, se voient ponctionner sur leur revenu commun 34 euros par mois, et non pas zéro euro chacun. Michel, ancien instituteur célibataire, perd 35 euros mensuels sur sa pension de 2 058 euros net, parce que ses retraites complémentaires lui font dépasser le plafond de 1 200 euros net. Sandrine perçoit 900 euros net de retraite par mois, plus 500 euros de pension de réversion de son mari décédé. Le montant total dépassant 1 200 euros, elle subit la hausse de la CSG.

ces amendements proposent de réduire de 1,7 point le taux de la CSG sur les pensions de retraite pour l'amener à 6,6 %, soit

ne me convient pas du tout, parce que cela veut dire que l'on entérine une baisse forte de pouvoir d'achat pour les retraités. Vous savez, les retraités savent compter,

Oui, madame la présidente, nous maintenons notre amendement, car cette proposition ne nous convient pas du tout. Les quelques exemples que j'ai cités dans mon intervention montrent à quel point les retraités vont perdre en pouvoir d'achat. Nous ne pouvons pas l'accepter. La parole

de trouver un prélèvement de 1 milliard d'euros sur les OCAM, les organismes complémentaires d'assurance maladie, et que nous avons assumé de proposer le recul de l'âge légal de la retraite.

demain la désindexation des retraites -allait avoir pour conséquence une baisse du pouvoir d'achat des retraités. D'ailleurs, ils expriment

des retraités et des citoyens qui ne sont pas forcément très satisfaits des mesures prises par le Gouvernement. Bien évidemment, la hausse de la CSG mécontente les retraités. Bien évidemment, la non-indexation ou la sous-indexation

dans l'intérêt de la sécurité sociale et dans l'intérêt du Sénat. Essayez de nous suivre, s'il vous plaît

Cet amendement vise à exonérer de CSG sur les revenus fonciers les retraités dont le revenu fiscal de référence ne dépasse pas 11 018 euros pour une personne seule et 16 902 euros pour un couple.

l'avis du Gouvernement ? Monsieur le sénateur, l'exonération que vous proposez porterait sur les seuls revenus fonciers perçus par certains pensionnés. Il nous semble qu'elle créerait des inégalités de traitement importantes au détriment des personnes modestes, qu'elles soient pensionnées ou non. Ainsi, si on imagine deux retraités dont le niveau de pension est le même et qui ont tous les deux un revenu fiscal de référence inférieur au seuil que vous avez fixé, seul celui qui aurait des revenus fonciers, disposant donc d'une source de revenus supplémentaires, serait avantagé par la suppression des prélèvements. Au-delà de cela, rien ne justifierait de ne pas tenir compte de ce critère de revenu fiscal de référence pour l'ensemble des redevables de la CSG et des prélèvements sociaux sur les revenus du capital, notamment les actifs. La mesure que vous proposez présente donc un risque juridique élevé. Par ailleurs, et je rejoins tout à fait M. le rapporteur général, une telle exonération porterait atteinte à l'universalité des prélèvements sociaux assis sur les revenus du capital, qui ont vocation à s'appliquer de la même manière à tous les redevables, indépendamment de leur niveau de ressources. À cet égard, les prélèvements sociaux

J'entends votre argument selon lequel la proposition vise à préserver les retraités modestes qui bénéficient d'un patrimoine foncier, notamment dans le secteur agricole. Il ne nous paraît cependant pas très efficace de chercher à répondre à la situation particulière des petites retraites agricoles par une réduction de la fiscalité du patrimoine,

évidemment à la disparition de la taxe d'habitation, à tout ce que nous faisons pour le reste à charge zéro ou l'aide à la complémentaire santé ... Autant de mesures en faveur des retraités les plus modestes. La CSG ne permettra pas de redistribuer du pouvoir d'achat

et le taux supérieur. Les retraités sont redevables sur leur pension suivant le niveau des revenus, selon des modalités différentes. Il est important de le rappeler. Ils ne paient rien en dessous de 11 018 euros de revenu fiscal de référence.

Désormais, il faudra dépasser le seuil de revenus pendant deux années consécutives pour se voir appliquer le taux maximal. Dans un souci de cohérence, la commission a estimé qu'il faudrait peut-être appliquer le même critère de dépassement du seuil de revenus de deux années de suite pour le passage du taux nul au taux intermédiaire, c'est-à-dire de 0 à 3,8 %. 0 à 3,8 %. C'est ce que nous proposons dans l'amendement n° 57. Cette disposition, qui concerne les revenus les plus modestes,

aménager la hausse de 1,7 point de la CSG pour les ménages dont le revenu fiscal de référence se situait juste au seuil et de façon intermittente. Elle visait à stabiliser les personnes assujetties lorsqu'elles dépassaient ce seuil deux années d'affilée. Le Gouvernement et le Premier ministre permettre à ces 300 000 foyers d'attendre deux années successives de dépassement du seuil pour être assujettis au taux majoré.

préexiste depuis des années. Votre proposition va bien au-delà d'une mesure de correction qui serait issue de la loi de financement de la sécurité sociale votée en 2018. Elle concernerait

Avec cet article 11, le Gouvernement propose de corriger les effets néfastes à la marge, pour certains Français modestes, de la hausse de la CSG de 1,7 point votée l'année dernière. Nous avions déjà dénoncé ces effets pervers qui ont eu des conséquences diverses sur le pouvoir d'achat des Français. Je pense d'abord aux fonctionnaires : le Gouvernement avait prévu une compensation à hauteur de 3 milliards d'euros, c'est-à-dire en dessous de la hausse de la CSG, ce qui s'est traduit par une perte de pouvoir d'achat. aux retraités : la hausse concernait celles et ceux qui sont actuellement assujettis au taux de 6,3 %. Ainsi, pour une personne seule, cette hausse s'applique dès que le revenu fiscal de référence dépasse soit 1 289 euros par mois si la personne a moins de 65 ans et 1 394 euros par mois si elle a plus de 65 et républicain a estimé qu'appliquer une telle hausse sans compensation aux retraités n'était pas acceptable en termes de pouvoir d'achat. Or le correctif proposé actuellement par le Gouvernement est insuffisant puisqu'il ne couvre que les hausses de CSG exceptionnelles, celles qui sont dues à des variations extraordinaires de revenu des foyers modestes- par exemple, la plus-value lors de la vente d'un bien. Ce rectificatif ne corrige ou très à la marge -la perte de pouvoir d'achat pour les Français modestes. Telles sont les raisons pour lesquelles, afin d'obtenir un équilibre entre le maintien du pouvoir d'achat des retraités français et l'exigence de sérieux dans la gestion des finances publiques, nous proposons d'introduire plus de progressivité dans le taux de la CSG. Nous proposons que la hausse de CSG pour les retraités ne s'applique pas pour les montants de retraite inférieurs au coût moyen d'une maison de retraite médicalisée. Nous proposons également que cette progressivité prenne en compte des seuils de revenus adaptés à la situation socioéconomique spécifique de la métropole, en premier lieu, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, en deuxième lieu, de

Il faut rappeler que, comme les auteurs ne cotisent pas au titre de l'assurance chômage, ils n'ont pas bénéficié des mesures de compensation de la hausse de la CSG. Ils ont donc subi une perte nette de revenus, à la différence du reste de la population. Lors des débats sur ce sujet, l'année dernière, le Gouvernement avait reconnu cet oubli et s'était engagé à prévoir un système permettant une compensation pérenne. Pour 2018, un décret a été pris le 15 mai dernier instituant une mesure de soutien au pouvoir d'achat des artistes auteurs ; 18 millions d'euros

suivantes. Le ministère de la culture et le ministère des affaires sociales ont reçu, le 21 juin dernier, l'ensemble des organisations d'artistes auteurs pour un échange autour de cette problématique,

d'alerter le Gouvernement sur la situation des artistes auteurs, qui ont vu leur pouvoir d'achat diminuer à la suite de la hausse de la CSG. Comme l'a rappelé Mme Morin-Desailly, les artistes auteurs n'ont pas bénéficié de mesures de compensation, puisqu'ils ne cotisent pas à l'assurance chômage. Le Gouvernement avait reconnu un oubli

compensant sur le long terme l'augmentation de la CSG. De surcroît- il est important de le souligner -, il ne concerne que les auteurs affiliés, et non l'ensemble des auteurs assujettis.

impossible qu'une catégorie de notre population- les artistes auteurs -ne puisse pas bénéficier, comme l'ensemble des actifs de notre pays, de la compensation de la hausse de la CSG. Je pense, madame la ministre, qu'il est vraiment temps

ont rappelé que, l'année dernière déjà, nous avions posé au Gouvernement la même question, et que nous attendions de sa part une réponse opérationnelle.

Pour l'année 2018, à titre transitoire, le Gouvernement a souhaité garantir une égalité de situation entre les artistes auteurs et les salariés en prévoyant une modalité de compensation adaptée à la situation spécifique de ces personnes. Une aide de l'État égale à 0,95 % du revenu artistique. Elle sera versée avant la fin de l'année 2018. Ce montant est à la hauteur de la perte de pouvoir d'achat issue de la hausse de la CSG. En 2019, le même dispositif sera reproduit, élargi à l'ensemble des artistes auteurs qui se feront connaître auprès des organismes agréés. Il n'est Il n'est en effet pas possible de mettre en oeuvre un dispositif pérenne dès 2019, comme vous le souhaitez, en raison du transfert de recouvrement des cotisations URSSAF, qui se fera en deux temps en 2019 et en 2020. En revanche, à partir de 2020, le Gouvernement a retenu une solution pérenne, à savoir la prise en charge d'une partie des cotisations vieillesse, afin de compenser la perte de pouvoir d'achat de manière individualisée et contemporaine à l'acquittement des prélèvements sociaux. La prise en charge budgétaire de cette compensation reviendrait à l'État, pour un montant annuel estimé à 18 millions d'euros.

Il prévoit le principe et la modalité de la prise en charge des cotisations retraite, tels que je viens de vous les exposer. Il est rédigé ; il sera publié avant la fin de l'année. L'objet de vos deux amendements, mesdames les sénatrices, est donc satisfait.

les artistes que nous voyons travailler sur l'ensemble de nos territoires. Nous pouvons vous faire confiance,

Madame la ministre, vous avez bien voulu apporter quelques éléments d'explication. Il n'en demeure pas moins qu'on constate, à juste titre, comme l'ont rappelé M. Brisson et

La situation est tout de même paradoxale : on se fait une fierté de nos auteurs, de nos écrivains, de nos artistes, on les revendique comme patrimoine de notre nation, dont ils participent au rayonnement, mais on ne prend pas les mesures adéquates en temps utile pour résoudre leurs problèmes particuliers. Il faut donc envoyer un signal fort pour résoudre définitivement ces questions. Nous comptons donc sur vous, madame la ministre, pour faire avancer définitivement ce dossier.

Jean-Marie Morisset. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a créé une taxe sur le chiffre d'affaires des distributeurs de tabac, afin de financer le fonds de lutte contre le tabagisme à hauteur de 130 millions d'euros par an. Cette taxe pose aujourd'hui d'importants problèmes de recouvrement qui mettent en péril le financement de la lutte contre le tabagisme, la répercussion de la taxe sur les fabricants de tabac étant actuellement source de nombreux contentieux juridiques. En effet, la taxe sur les distributeurs de tabac ne concerne qu'un seul acteur économique majeur la société Logista, qui assure la distribution de la quasi-totalité des produits de tabac en France. Cette société est actuellement en péril, ne pouvant assumer seule cette charge fiscale qui devrait peser directement sur les fabricants de tabac. C'est la raison pour laquelle le présent amendement vise à réintégrer la taxe sur les distributeurs dans les droits d'accises sur les produits de tabac, par une augmentation à due concurrence de la part spécifique de ces droits. En éliminant le risque contentieux et en faisant supporter le paiement de la fiscalité par les fabricants de tabac, et non plus par les distributeurs, la mesure proposée garantit les moyens dédiés à la lutte contre le tabagisme, dans le cadre du nouveau fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives créé à l'article 38 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale.

constitue une ressource précieuse pour alimenter le fonds de lutte contre le tabagisme, qui sera bientôt élargi aux addictions liées à toutes les substances psychoactives. Par ailleurs, remplacer cette contribution par un relèvement des droits d'accises ne garantit pas une taxation des fabricants, puisque ces droits sont exigibles des fournisseurs à la mise en consommation ou à l'importation.

aux prélèvements sociaux : contribution sociale généralisée, contribution au remboursement de la dette sociale, prélèvement social, contribution additionnelle et prélèvement de solidarité. Toutefois, l'affaire des « CumEx Files », révélée par une dizaine de médias le mois dernier, a démontré la gigantesque évasion fiscale dont sont victimes des États européens, parmi lesquels l'Allemagne, le Danemark et la France, pour un préjudice estimé à plus de 55 milliards d'euros. Une bande de, de banques et d'avocats a mis en place un système pour frauder le fisc allemand. Exploitant une faille de la loi, ils se sont en effet échangé de gros volumes d'actions, au moment précis où le dividende était versé aux actionnaires, afin de brouiller l'identité des véritables bénéficiaires de ces titres. Cette affaire a mis au jour des montages financiers sur les dividendes qui permettent de douter de la réalité de l'efficacité des systèmes existants. C'est la raison pour laquelle nous proposons de mettre à contribution les revenus financiers afin de dégager de nouvelles recettes pour financer la protection sociale. À rebours des politiques d'exonérations de cotisations patronales- nous avons déjà expliqué à plusieurs reprises qu'elles endettent la sécurité sociale -, nous proposons de soumettre à cotisations sociales les dividendes Je rappelle que le montant des dividendes versés par les entreprises françaises en 2018 a été de 51 milliards d'euros, soit le montant le plus important d'Europe. chers collègues, de mettre à contribution les revenus financiers des sociétés financières et non financières, afin d'inciter l'embauche et l'investissement. Voilà une proposition qui, je l'espère, vous séduira ! Quel est l'avis de la commission ? Ces revenus

âgées en perte d'autonomie, est à bout de souffle. Si, sur le principe, notre groupe a toujours été opposé à la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie, la CASA, c'est que nous estimons que ce n'est pas aux seuls retraités de payer pour leur autonomie. De l'argent, il y en a ; il suffit de se donner les moyens d'aller le chercher ! Par cet amendement, nous réclamons donc la création, en miroir de la CASA actuelle, d'une contribution de solidarité des actionnaires, prélevée sur les dividendes perçus à hauteur de 2 %. Cette contribution permettrait d'abonder les comptes de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie d'un montant proche de 1 milliard d'euros. Cette somme permettrait d'assurer une revalorisation des tarifs de l'aide à domicile jusqu'à approcher 25 euros de l'heure. Ces structures traversent une véritable situation de crise ; elles nous appellent au secours

a précisément pour mandat de proposer de nouvelles pistes de financement plus structurelles. Attendons ! La commission a donc émis un avis défavorable

sur l'évolution de notre modèle de prise en charge de la perte d'autonomie, avec un volet sociétal, mais aussi, évidemment, un volet financier. Nous ne souhaitons donc pas engager la moindre réforme du financement de la dépendance avant le projet de loi qui sera déposé sur ce

s'appliquant aux assurances santé à but lucratif. Nous proposons de taxer celles-ci à hauteur de 20 % de leurs bénéfices annuels. Le produit de cette taxe sera affecté à la branche maladie des comptes de la sécurité sociale. la DREES, a publié son bilan sur l'ouverture depuis le 1 janvier 2016 du marché des complémentaires de santé aux assureurs privés lucratifs : ce document montre que cette ouverture du marché a largement bénéficié aux assureurs privés au détriment des mutuelles. Ainsi, parmi les neuf organismes qui ont accru leurs parts de marché entre 2015 et 2016, cinq sont des assureurs et quatre des institutions de prévoyance. Huit de ces groupes étaient déjà des acteurs majeurs des complémentaires et ont donc conforté leurs positions, contrairement aux acteurs mutualistes. Depuis l'ouverture du marché, ces organismes ont dégagé 900 millions d'euros supplémentaires- j'insiste sur ce montant. Les organismes mutualistes ont, eux, souffert de la mesure, puisqu'ils perdent des parts de marché. Or ils exercent

En effet, la santé n'est pas et ne doit pas être considérée comme un bien marchand. Il appartient à l'État d'exercer un contrôle sur les activités des assureurs privés, afin d'être sûr que leur priorité reste la santé de leurs assurés et non la seule augmentation de leurs bénéfices. Pour cette raison, nous proposons la création de cette taxe additionnelle, qui permettra d'apporter d'importantes recettes à la sécurité sociale, lesquelles pourront être affectées à la branche maladie, toujours déficitaire. Quel est l'avis de la commission ? Cet amendement ? Cet amendement vise à instaurer une taxe de 20 % sur le bénéfice des sociétés d'assurance au profit de la branche maladie.

à exonérer les hôpitaux publics du versement de la taxe sur les salaires, afin de leur permettre de dégager des ressources supplémentaires. Toutefois, les financements publics dont bénéficient les hôpitaux intègrent d'ores et déjà la dépense que représente cette taxe. On parle ainsi d'un effet circulaire

En réalité, dans sa réponse au référé de la Cour des comptes sur ce sujet, cette année, le Premier ministre a même confirmé qu'« une diminution à due concurrence des subventions et dotations publiques octroyées aux employeurs concernés devrait être opérée

! Par ailleurs, comme nous l'avons évoqué en commission, un risque de rupture d'égalité devant les charges publiques existe, pas seulement entre établissements publics et établissements privés à but non lucratif, mais aussi entre certains établissements de santé privés à but lucratif qui paient la taxe sur les salaires, dans la mesure où toutes les activités de dispensation des soins sont exonérées de TVA. Par conséquent, comprenez que nous ne soyons guère enthousiastes

créerait une différence de traitement entre les établissements publics de santé qui seraient exonérés de la taxe sur les salaires, alors que les établissements privés à but non lucratif demeuraient, eux, assujettis à la même taxe. Il y a bien un défaut de rédaction. Au-delà, cette

est une contribution à la charge des employeurs pesant sur des éléments de rémunération alternatifs au salaire et non soumis à cotisations sociales, c'est-à-dire principalement l'intéressement, la participation, l'actionnariat salarié.

du forfait social, madame la ministre. En effet, il exonère du forfait social les entreprises de moins de 50 salariés pour leurs versements liés aux dispositifs de participation financière, ainsi que les entreprises entre 50 et 250 salariés pour leur versement au titre de l'intéressement.

aménage aussi un nouveau taux dérogatoire de forfait social à 10 % pour l'ensemble des entreprises, lorsque celles-ci versent des sommes à leurs salariés au titre de l'actionnariat salarié.

? D'ailleurs, je ne suis pas convaincu que le forfait social soit le seul frein à la mise en place des accords de participation. Faute d'avoir pu mener à bien une telle réflexion,

à aligner la nouvelle dérogation concernant l'actionnariat salarié sur le taux dérogatoire de 8 %, afin de ne pas créer un quatrième taux dérogatoire. Madame la ministre, j'espère que vous serez sensible au souci du Sénat de ne pas trop complexifier le dispositif, tout en comprenant qu'un taux de 20 % puisse être un frein pour les PME dans le développement de l'épargne ou de l'actionnariat salarié.

avec des mesures fortes : la suppression du forfait social sur les versements des primes d'intéressement pour les entreprises de moins de 250 salariés et la suppression de ce même forfait sur les versements liés aux primes de participation, ainsi que sur les abondements des employeurs pour les entreprises de moins de 50 salariés. Pour diffuser plus largement l'actionnariat salarié, le Gouvernement a également souhaité diviser par deux le taux de forfait social qui s'applique au versement de l'employeur dans le cadre de ces plans. Celui-ci est donc fixé désormais à 10 % pour toutes les entreprises. Si ce taux est ramené à 8 %, cet abaissement supplémentaire entraînerait une perte de recettes pour la sécurité sociale d'environ 10 millions d'euros. Il conduirait aussi à placer le taux de prélèvement sur ces formes de rémunération au même niveau que celui qui concerne les contributions des employeurs au financement des dispositifs de prévoyance. Or ces derniers doivent conserver un caractère incitatif au moins équivalent à celui de l'abondement de l'employeur, afin de permettre une couverture de qualité pour les salariés. Nous souhaitons qu'un différentiel

en rétablissant à hauteur de 30 % le taux de la contribution sur ces actions. Le dispositif permettant la distribution d'actions gratuites pour la participation salariale avait été inscrit dans la loi Macron de 2015. Il avait pour objectif de permettre à un créateur d'entreprise n'ayant pas les moyens de recruter un ingénieur, pour ne pour ne prendre que cet exemple, d'attribuer à ce dernier des actions gratuites, afin de l'intéresser au développement de la société. Initialement, l'esprit ayant présidé à la création de ce mécanisme était de permettre aux petites entreprises d'être plus attractives pour les salariés.

qu'elles peuvent parfaitement mettre en oeuvre, afin d'attirer les salariés, sans avoir besoin de bénéficier d'un allégement de contribution, contrairement aux petites et moyennes entreprises. C'est pourquoi, dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2016, un taux de 30 % a été fixé pour les grandes entreprises, tandis qu'un taux zéro était appliqué aux PME. Cette disposition se justifiait parfaitement, puisqu'elle permettait un traitement différencié selon la taille, donc selon

payée par les complémentaires, avec un rendement de 300 millions d'euros. Le forfait patientèle est issu de la convention du 6 décembre 2016 conclue entre les syndicats médicaux, les complémentaires santé et l'assurance maladie, qui prévoit de valoriser les modes de rémunération alternatifs à l'acte des médecins traitants. Le nouveau forfait intitulé « forfait patientèle médecin traitant » prévoit de revaloriser le financement des actes du médecin traitant dont la patientèle répond à certaines caractéristiques d'âge, de pathologie et de précarité. Ainsi les médecins disposant d'une patientèle en ALD, affection longue durée, ou post-ALD, d'une patientèle bénéficiaire de la CMU-C et d'une patientèle âgée voient leurs actes majorés. En contrepartie du financement au forfait, les médecins s'engagent à ne pas pratiquer de dépassements d'honoraires. De leur côté, les organismes complémentaires d'assurance maladie sont mis à contribution pour ce qui concerne le financement des rémunérations forfaitaires des médecins traitants à hauteur de 150 millions d'euros en 2017, 250 millions d'euros en 2018 et 300 millions d'euros l'an prochain. La contribution transitoire à l'origine des complémentaires est transformée avec l'article 12 en une taxe de 0,8 % qui finance les forfaits des médecins. Si nous refusons cette transformation, c'est, d'une part, d'une part, parce qu'elle transfère le financement de la sécurité sociale vers les complémentaires santé, d'autre part, parce que le paiement de cette taxe sera inévitablement acquitté par les assurés sociaux pour lesquels les cotisations mutualistes seront revues à la hausse. Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article. Quel est l'avis de la commission ?

trahir sa parole. Quel est l'avis du Gouvernement ? Madame la sénatrice, vous rappelez que nous avons, par la voie conventionnelle, stabilisé la participation des organismes complémentaires aux nouveaux modes de rémunération des médecins-

cet amendement supprimerait totalement la participation des organismes complémentaires au financement du forfait patientèle des médecins traitants. C'est totalement contraire à la philosophie des réformes que nous menons. C'est la raison

La contribution actuellement prévue est assise sur les sommes entrant dans le champ de la taxe de solidarité additionnelle, à savoir le montant des primes et cotisations d'assurance maladie complémentaire des OCAM, mais également les garanties assurant le versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale qui relèvent en pratique des contrats de prévoyance. Or la contribution prévue à l'article 12 ne concerne que les frais de santé : elle a vocation à permettre la prise en charge d'une prestation de soins. C'est pourquoi il serait plus cohérent d'en exclure les contrats de prévoyance. Toutefois, afin de conserver le rendement de 300 millions d'euros souhaité par le Gouvernement, le taux de la contribution serait fixé à 0,83 % au lieu des 0,8 % prévus initialement.

Cet amendement vise à sécuriser dans le temps la participation des organismes complémentaires santé au financement des nouveaux modes de rémunération. L'article 12, dans sa rédaction qui est issue des débats à l'Assemblée nationale, prévoit de supprimer la participation des organismes complémentaires au financement du forfait patientèle des médecins traitants à l'échéance de la convention médicale, en 2021. Je rappelle que cette taxe, d'un montant d'environ 300 millions d'euros, a été instituée en concertation avec les organismes complémentaires, en raison de l'impossibilité pour eux de financer directement les médecins qui perçoivent ce forfait. Le lien fait avec la convention médicale est logique, mais la façon dont cet article l'exprime est de nature à soulever des difficultés juridiques, en particulier en ce qu'il remet en cause le plein exercice par le législateur de la compétence en matière fiscale qui lui est conférée par l'article 34 de la Constitution. l'amendement vise à ne plus renvoyer à une situation conventionnelle les conditions d'application de cette imposition. Il tend à stabiliser le principe de la taxe jusqu'à l'année d'expiration de la convention, en 2021, et à maintenir le lien logique avec la convention médicale, tout en renvoyant à un acte législatif exprès l'abrogation de la taxe, ce qui semble plus conforme à la hiérarchie des normes. Il s'agit par ailleurs de procéder à une précision rédactionnelle quant à l'assiette de la taxe, afin d'éviter toute ambiguïté. L'assiette de la contribution sera bien alignée sur celle de la TSA. Sont donc explicitement exclues les garanties qui sont déjà exonérées de la TSA, par exemple les garanties d'indemnités journalières complémentaires des contrats agricoles.

sécuriser les modalités prévues par l'Assemblée nationale pour limiter l'application de ce dispositif fiscal aux seules années d'application de la convention médicale

Le 13 juin 2016, l'association médicale de solidarité internationale Médecins du monde dénonçait dans une campagne-choc les bénéfices exorbitants des laboratoires pharmaceutiques.

entre en contradiction avec la mission d'intérêt général visant à mettre à disposition les traitements nécessaires aux patients. Il est

selon le recours ou non, par les assurés, à des professionnels partenaires d'un réseau de soins. La mise en place de cette réforme va recentrer ces réseaux sur les offres du marché libre pour lesquelles les remboursements de l'assurance maladie obligatoire seront, pour ce qui concerne l'optique notamment, fortement diminués. Dans ce cadre, cet amendement tend à éviter qu'à l'occasion de ces évolutions, les assurés ne puissent se voir appliquer des remboursements différenciés par leur organisme complémentaire. Les contrats qui prévoiraient des clauses de ce type ne seraient pas éligibles au taux réduit de taxe de solidarité additionnelle, ou TSA, applicable aux contrats responsables et solidaires.

des contrats responsables, un remboursement différencié. Dans les faits, cette pratique leur permet de moins bien rembourser leurs assurés qui ne se rendraient pas chez un professionnel de santé affilié à leur réseau de soins, y compris lorsqu'il s'agit de leur professionnel de santé habituel. Alors que de nombreux territoires ne disposent pas de professionnels de santé affiliés à un tel réseau, le remboursement différencié pourrait aggraver les inégalités territoriales d'accès aux soins.

de la réforme du reste à charge zéro, qui va recentrer les réseaux de soins sur le marché libre, il peut être utile d'éviter le développement de telles pratiques de différenciation des prises en charge. Sans être le seul levier pour inciter les assurés à recourir aux professionnels partenaires du réseau, le remboursement différencié serait le fait, d'après un récent rapport de l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales, d'environ un tiers des organismes. Forte de tous ces arguments, la commission a émis un avis favorable sur ces quatre amendements

Vous proposez de majorer le taux de TSA pour les contrats responsables permettant un remboursement différencié en fonction du choix de l'assuré.

aux collectivités territoriales, notamment aux plus petites d'entre elles- communes, syndicats intercommunaux -de recourir à un dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement des cotisations et des contributions sociales. L'article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoit que les dispositifs du titre emploi service entreprise et du chèque emploi associatif soient ouverts à compter du 1 janvier 2019 à toutes les entreprises et associations quelle que soit leur taille, et non plus aux seules structures de moins de vingt salariés. C'est pourquoi, pourquoi, en toute logique, dans un souci de simplification du fonctionnement des collectivités territoriales ou de leurs groupements, il nous paraît pertinent de permettre à ceux-ci d'accéder à ces dispositifs, au même titre que les associations ou les entreprises.

afin d'attendre que le territoire soit entièrement câblé et que tout le monde puisse avoir accès à la précieuse fibre. Quel est l'avis de la commission ? La ? La commission soutient, bien sûr, le renforcement des obligations de dématérialisation, mais il ne faut pas entraver le développement des travailleurs indépendants sur le territoire,

La commission ne dispose pas d'informations suffisamment précises sur la situation des travailleurs indépendants outre-mer et sur leur accès à internet. C'est pourquoi elle a souhaité se

vous soulignez le problème des zones blanches. En réalité, dans les outre-mer, comme partout, d'ailleurs, les travailleurs indépendants, quel que soit leur lieu d'exercice, zone blanche ou pas, effectuent déjà par voie dématérialisée leurs déclarations à l'administration fiscale

et simultanée au paiement des cotisations et du prélèvement à la source sur le salaire du salarié. L'employeur n'a donc plus qu'à faire une déclaration par mois au CESU, qui se charge ensuite de toutes les formalités, y compris le prélèvement du salaire pour le reverser au salarié. Ce service permet également au particulier de bénéficier des aides auxquelles il a droit pour l'emploi de ce salarié, en particulier le complément de libre choix du mode de garde, le CMG. peut donc en bénéficier concomitamment au versement du salaire, ce qui représente un avantage en trésorerie intéressant pour les particuliers. Il s'agit donc d'un service particulièrement innovant, qui simplifiera la vie des particuliers-employeurs. Le recours à ce service est conditionné à l'accord du salarié pour que son salaire soit versé après retenue du prélèvement à la source des cotisations par l'intermédiaire du centre CESU et du centre Pajemploi, lesquels auront prélevé les sommes nécessaires sur le compte de l'employeur. En outre, selon la loi, le particulier-employeur qui demande à adhérer à ce service doit transmettre la copie de l'accord écrit de son salarié au centre CESU et à Pajemploi. Cette formalité supplémentaire risque cependant de complexifier fortement l'adhésion et l'utilisation du service. Il vous est donc proposé de supprimer l'obligation de transmettre ce justificatif, afin de permettre une adhésion plus simple et plus rapide. Une telle telle évolution ne dispense évidemment pas l'employeur de l'obligation d'obtenir l'accord de son salarié. Mais, au lieu de la transmission du justificatif, le Gouvernement propose que les organismes mettent en place un système d'information avertissant immédiatement un salarié de l'adhésion de son employeur au service, afin de s'assurer que les deux parties sont pleinement d'accord. L'adoption de cet amendement permettrait donc à la fois de simplifier les démarches de l'employeur et de préserver les droits du salarié.

l'essentiel de mes amendements portaient justement sur ces zones blanches, où il n'y a vraiment pas de réseau. Hier, lors de la

qui a intentionnellement fourni à un cotisant une prestation ayant directement contribué à la commission des actes constitutifs de l'abus de droit en cause ou à la dissimulation de ces actes est redevable d'une amende. telle disposition pose deux problèmes. Premièrement, il faut informer lesdits professionnels de la possibilité de saisir le comité des abus de droit, qui donne un avis.

D'une part, au fil des années, le législateur a banalisé le travail dissimulé, à tel point que beaucoup le pratiquent sans le savoir. Ainsi en est-il du cas du client de bar qui vient rapporter son verre au comptoir, de l'entraide entre voisins, de la personne qui vient aider son frère sur un marché, des laissés-pour-compte qui reçoivent un modeste pécule d'une communauté d'Emmaüs, de l'entraide familiale, etc. D'autre part, les sanctions constituent un « arsenal d'une violence juridique et économique inouïe Afin que les décisions prises soient réfléchies, nous proposons que le procès-verbal soit contresigné par le directeur de l'organisme effectuant le recouvrement. Non seulement cette solution semble évidente s'agissant d'une décision grave, mais on notera de surcroît que le contreseing est déjà prévu pour des situations de moindre gravité, comme l'absence de bonne foi du cotisant.

D'une part, un agent constate les infractions et en informe la personne contrôlée. D'autre part, le directeur de l'organisme s'assure du recouvrement des sommes dues et dispose de prérogatives, dont la prise de mesures conservatoires. Ces deux actions sont complémentaires, mais elles sont distinctes. Elles sont assurées dans le cadre d'un échange avec la personne contrôlée, d'autant que cette dernière peut toujours saisir la commission de recours amiable en cas de difficulté.

Aujourd'hui, lorsque la mission nationale de contrôle, la MNC, annule une décision de la commission de recours amiable, le cotisant est seulement informé du rejet de son recours.

contrôle, la dernière notification assurée au cotisant précise : la délibération initiale de la CRA ; le motif d'annulation de la délibération retenu par la MNC ; la nouvelle décision de la CRA au regard de la position de la MNC. Cette disposition vise à informer précisément le cotisant des raisons ayant motivé le refus de son recours. Or il est possible de constater que ce principe n'est pas appliqué.

commission ? Il est effectivement souhaitable d'accroître l'information du cotisant sur l'annulation d'une décision de la commission de recours amiable le concernant et sur les motifs ayant conduit à cette annulation. La commission émet donc un avis favorable Quel est l'avis du Gouvernement ? Il est proposé d'introduire le droit pour le cotisant de connaître le motif du refus de la mission nationale de contrôle à la suite d'une décision prise par une caisse. À nos yeux, il n'y a pas d'intérêt à informer le cotisant de l'intervention de la mission nationale de contrôle, qui exerce un contrôle de légalité préalable, c'est-à-dire un acte préparatoire à une décision finale, puisque la décision n'est pas encore intervenue.

Cet amendement prévoit la création d'un interlocuteur qui pourrait être saisi par le cotisant « en cas de difficultés rencontrées au cours de la vérification ». Aujourd'hui, dans l'hypothèse d'un contrôle, le cotisant est seul face à l'inspecteur. Certes, une procédure contradictoire a été retenue, mais elle se déroule devant le même inspecteur, qui changera rarement d'avis. Il serait donc judicieux de créer les conditions d'un véritable dialogue. Quel est l'avis de la commission ? Cet amendement

cet amendement est prévue la possibilité de prolonger la procédure contradictoire. En effet, il est illusoire, surtout pour les entreprises assez importantes, de pouvoir répondre à des observations de l'URSSAF en trente jours.

Or un tel droit, qui correspond d'ailleurs assez bien à certaines pratiques, est envisageable sans risque pour les finances publiques. En effet, depuis l'année dernière, les délais de prescription des créances sont suspendus pendant la période contradictoire, ce qui permet de dégager davantage de temps pour que des échanges d'arguments puissent se tenir sans prendre de risques pour le recouvrement des sommes dues.

C'est pourquoi les personnes ayant recours à des montages relevant de l'abus de droit, ainsi que celles qui recourent au travail dissimulé ou à la dissimulation d'activité sont exclues de cette mesure favorable. C'est d'ailleurs la règle qui prévaut en matière fiscale et dont les auteurs de

Il serait souhaitable de mettre fin à un imbroglio juridique en matière de recouvrement des cotisations. En effet, une URSSAF, afin d'accélérer la procédure, est-elle en droit de décerner une contrainte, dans le cadre du contentieux du recouvrement, en cas de saisine préalable de la commission de recours amiable par le débiteur, laquelle relève du contentieux général ? La réponse paraissait négative. Toutefois, faute de texte, la Cour de cassation a décidé l'inverse, obligeant ainsi le débiteur à mener deux actions de front. Il convient donc de mettre fin à cette étrangeté.

En effet, prévoir dans les dispositions générales du contentieux la suspension de toute procédure de recouvrement en cas de contestation nous paraît risqué.

des audiences et de l'engorgement des juridictions, avec une telle mesure, le recouvrement des cotisations pourrait prendre jusqu'à cinq ans à dix ans. Le risque pour les URSSAF serait important. Le montant total des redressements effectués par les URSSAF l'année dernière était de 1,3 milliard d'euros. Cet amendement, en allongeant considérablement les délais, nous mettrait quelque peu en difficulté

Mme Pascale Gruny. Il convient de rappeler que, dans tous les cas, le cotisant doit avoir la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec l'inspecteur du recouvrement sous peine d'irrégularité de la procédure de contrôle. Il s'agit ici d'un rappel solennel qui doit, dans l'intérêt des parties, être clairement inscrit dans les textes. Quel est l'avis de la commission ?

Par ailleurs, le caractère contradictoire de la procédure de contrôle est strictement garanti par les textes, notamment par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et par d'autres articles qui reprennent les garanties fixées par le juge. Il existe donc un encadrement assez strict du contrôle

Il ne sera même pas possible de savoir si l'absence d'échange oral pendant le contrôle est liée à une contrainte d'organisation des travaux lors du contrôle, à un choix de la personne contrôlée ou à un tout autre facteur. Voilà pourquoi je vous propose d'en rester là et

En effet, à l'issue d'un contrôle, l'agent chargé de ce dernier adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure. Dans le cas d'une vérification, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire. Toutefois, il n'est pas indiqué pendant combien de temps ce délai est suspendu : un mois, douze mois, cinq ans ? Cela ne contribue ni à la transparence ni à la sécurité juridique. Une entreprise contrôlée est en droit de recevoir les résultats du contrôle dans un délai raisonnable, d'autant que les majorations de retard courent pendant cette période. Pourtant, la disposition introduite par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 ne va pas dans ce sens et n'incite guère les organismes à « presser le mouvement », puisque toute la période depuis les observations jusqu'à la mise en demeure est suspendue. Or, justement, la loi est là pour prévenir les abus. Il est raisonnable de prévoir que le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard soit suspendu pendant la période contradictoire et pour une durée maximale de six mois. Quel est l'avis de la commission ? Le délai de Le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire.

est à Mme Pascale Gruny. Dans le cadre du travail dissimulé, les agents habilités à constater l'infraction peuvent procéder à des auditions. Toutefois, il n'est pas prévu qu'une copie du procès-verbal d'audition soit transmise au contrevenant. Cette situation ne garantit pas une procédure contradictoire, d'autant que, récemment, la loi pour un État au service d'une société de confiance, dans son article 39, a modifié le code de l'environnement prévoir la transmission obligatoire du procès-verbal au contrevenant. Quel est l'avis de la commission ? Le code du travail prévoit que les agents de contrôle du travail illégal peuvent procéder à l'audition d'une personne suspectée d'avoir commis une infraction. Certaines garanties du code de procédure pénale s'appliquent. Or ces règles ne comprennent pas la transmission du procès-verbal à l'auditionné. L'adoption de votre amendement, madame Gruny, créerait une importante dérogation à la procédure pénale, ce qui n'est pas souhaitable.

s'effectue « sauf instruction contraire du procureur de la République ». On peut donc conclure positivement que ce document peut être transmis. Or une telle garantie n'est pas apportée dans cet amendement.

Que reste-t-il de compétences aux parlementaires que nous sommes lorsque le code de la sécurité sociale dispose qu'un amendement est irrecevable

acceptable ! Je ne fais de procès à personne puisqu'il s'agit de la stricte application de la loi, confortée par le règlement du Sénat. Pour autant, quand pourrons-nous assumer notre fonction pour tenter d'améliorer l'organisation sanitaire, l'accès aux soins, etc. ? un hypothétique projet de loi sur la santé. Hormis cela, nous ne pouvons rien changer à l'organisation des soins ! Il conviendrait sans doute que nous y réfléchissions pour que chacun d'entre nous puisse avoir les moyens d'honorer les missions que la Nation lui confie

Mme Laurence Cohen. Le Gouvernement entend, avec l'article 15 et les mécanismes de sauvegarde applicables aux médicaments, substituer aux taux Lv et Lh un taux unique, le taux M. ferai pas de remarque particulière sur ce changement, si ce n'est qu'il s'agit de la troisième modification en la matière depuis 2015. Mais, et c'est ce sur quoi repose notre amendement, l'article 15 fixe le montant du taux M à 1,005 fois l'assiette de 2018, conformément aux engagements pris en juillet dernier lors du conseil stratégique des industries de santé. Concrètement, cela signifie que le chiffre d'affaires des industries considérées pourra donc progresser de 0,5 % sans que la clause M soit déclenchée.

comparé au taux de 0,3 % de revalorisation des prestations sociales, nous paraît quelque peu incongru, pour ne pas dire indécent. Nous proposons donc de limiter cette hausse à 0,3 % à l'instar de ce que prévoit généreusement le Gouvernement pour les prestations sociales : cela nous semble être une question d'équité. Vous remarquerez que nous tenons compte toutefois de la croissance de l'évolution du marché du médicament avec cette progression à 0,3 % pour, par exemple, prendre en considération l'arrivée sur le marché de médicaments innovants.

Pour cela, nous avons trois outils de régulation. D'abord, une action sur les volumes, car les Français consomment trop de médicaments, ce qui pose des problèmes de santé publique et de iatrogénie.

C'est un effort substantiel. Nous considérons qu'il faut trouver le bon équilibre. Dans le cadre du CSIS, a été votée une augmentation de 0,5 % du chiffre d'affaires. Nous nous sommes engagés sur ce point. Cela ne nous empêchera pas de réaliser le milliard d'économies

sur trois ans. Les baisses de prix et la pression économique, supérieure aux années antérieures, exercée en 2019 sur le médicament vont confisquer la part de croissance accordée par le taux de 0,5 %. Ce sont 1,8 milliard d'euros d'économies, soit la moitié des économies réalisées en matière de santé, alors que le médicament pèse 15 % des dépenses de l'assurance maladie. Les innovations seraient favorisées en augmentant raisonnablement ce taux à 1 %, ce qui, avec un ONDAM à 2,5 %, resterait soutenable et cohérent par rapport aux engagements pris lors du CSIS, d'autant que le Gouvernement possède des garanties pour que le marché ne s'envole pas avec la clause de sauvegarde et la baisse des prix. Ce taux de 1 % enverrait un message positif aux industries de santé, permettant ainsi la restauration d'une France attractive pour les investissements dans le domaine de la santé et l'accès aux médicaments pour les patients. Quel est l'avis de la commission ? Nous devons

sur les évolutions à attendre au cours des prochains exercices budgétaires, car la mesure n° 13 du CSIS prévoit que, pour améliorer la prévisibilité et la stabilité de la régulation, les paramètres de la clause de sauvegarde seront annoncés plusieurs années à l'avance.

ont été discutés longuement avec les industriels, puisque nous nous étions engagés à donner un peu plus de visibilité à la politique française en matière de médicaments. En tout état de cause, la clause de sauvegarde est un outil qui nous permet de

Les entreprises de répartition pharmaceutique disposent d'un large référencement des médicaments génériques destinés à l'approvisionnement des officines. Acteurs responsables, les grossistes-répartiteurs vont au-delà de leurs obligations légales sur ce segment qui ne leur imposent de disposer que du que du princeps et d'un générique. Ce faisant, ils constituent un levier puissant de développement du générique en France. Ils contribuent pleinement au développement de ce marché, en proposant l'ensemble des références génériques aux patients qui peuvent conserver leurs habitudes de traitement. Ils participent à la maitrise des dépenses de santé. Ils accompagneront le Gouvernement dans son objectif de renforcement de la substitution des princeps par les génériques. Or, dans son rapport annuel de 2017 sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, la Cour des comptes confirme la situation économique préoccupante des entreprises de la répartition

La situation est telle que les conditions dans lesquelles les répartiteurs distribuent ces médicaments ne sont pas économiquement supportables. Une concertation s'est d'ailleurs engagée sur le sujet avec la direction de la sécurité sociale, la DSS, mais les premiers éléments ne sont pas concluants, puisque l'application des projections conduirait à dégrader plus encore la situation présent amendement vise à retirer le segment des génériques de l'assiette de la taxe sur le chiffre d'affaires des distributeurs en gros et à pérenniser, ainsi, l'activité des grossistes-répartiteurs. Cette mesure, salutaire au regard de l'urgence, constituerait, par ailleurs, une mise en cohérence avec le cadre fiscal existant, les génériques étant déjà exclus d'une des trois composantes de cette taxe. Dans l'attente d'une refonte plus globale de la rémunération des grossistes-répartiteurs, cet amendement tend à instaurer une mesure d'urgence : l'exclusion des médicaments génériques de l'assiette de la taxe sur le chiffre d'affaires des distributeurs en gros.

vous avez déclaré dernièrement que la profession dont nous parlons, à savoir celle des répartiteurs, est très utile à la distribution des médicaments. Chacun le sait, la répartition joue un rôle majeur dans la chaîne du médicament : les entreprises de la répartition sont le lien essentiel entre l'industrie

une sécurisation des produits, un recyclage des médicaments, ainsi que la distribution de 75 % des médicaments génériques. Madame la ministre, vous avez indiqué souhaiter mettre en place une convention entre les médecins et les pharmaciens qui veulent voir augmenter le nombre de génériques. Pour autant, les territoires isolés ont besoin des grossistes-répartiteurs : il importe de continuer la livraison de médicaments de façon équitable sur l'ensemble de nos territoires. Nous avons donc intérêt à garder ce modèle économique efficace. Il est par conséquent essentiel de mettre en place cette mesure

Ces entreprises remplissent une mission essentielle pour nos concitoyens et nos territoires en permettant l'approvisionnement en médicaments de toutes les pharmacies de France, indépendamment du lieu d'implantation Dans ce secteur, des acteurs privés répondent à des obligations de service public- livraison des 22 0000 officines françaises dans un délai maximal de vingt-quatre heures après chaque commande, référencement d'au moins neuf médicaments sur dix et gestion d'un stock correspondant à au moins deux semaines de consommation -en contrepartie d'un encadrement de leur mode de rémunération par l'État. Or, dans son rapport annuel de 2017 sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, la Cour des comptes a confirmé la situation économique préoccupante des entreprises de la répartition. En effet, ce modèle hybride est aujourd'hui gravement fragilisé, ses missions n'étant plus suffisamment financées. En dépit de la concertation que vous avez engagée, madame la ministre, le secteur demande des mesures urgentes sans lesquelles l'approvisionnement quotidien des Français en médicaments pourrait être remis en cause, en particulier dans les territoires les plus fragiles où l'accès aux soins est souvent déjà difficile.

la suppression de la taxe sur le chiffre d'affaires des distributeurs en gros qui représente près de 20 % de leur marge, prévue à l'amendement n° 442 rectifié ; la réduction à 1 contre 1,75 % du taux de la première part de la taxe assise sur le chiffre d'affaires et prélevée par l'ACOSS au titre de la vente en gros de médicaments, prévue à l'amendement n° 445 rectifié. Ces mesures ont toutefois vocation à être transitoires en attendant que la concertation engagée avec les services ministériels aboutisse à une solution soutenable pour les entreprises de la répartition pharmaceutique, dans l'optique de garantir la pérennité de l'approvisionnement en médicaments de l'ensemble des citoyens et des territoires. Quel

Les difficultés s'expliquent notamment par le fait que leur rémunération est principalement assise sur le prix des médicaments livrés.

Après un examen attentif de cette question, je pense que l'exclusion des médicaments génériques de l'assiette de la taxe considérée ne constitue pas une solution pertinente et cohérente. Nous venons en effet, à l'article 15, de réintégrer ces médicaments dans l'assiette du montant M

40 millions d'euros aux grossistes-répartiteurs. Celle que je vous proposerai de retenir leur rapportera environ 30 millions d'euros. D'après ce que m'a indiqué la profession, cela lui permettra de garder la tête hors de l'eau en attendant une véritable réforme de son modèle économique. plat- je me tourne vers vous, madame la ministre -de la répartition pharmaceutique. La Cour des comptes, qui s'est penchée sur ce sujet, a recommandé la mise en place d'une rémunération en fonction des volumes de vente plutôt qu'en fonction des prix de vente. Je pense que c'est en effet la solution à mettre en oeuvre. Les grossistes-répartiteurs m'indiquent cependant qu'ils n'ont été reçus qu'une seule fois par vos services, madame la ministre, et que la réforme un temps envisagée est aujourd'hui au point mort. Pouvez-vous nous fournir quelques éclaircissements sur vos intentions, ainsi que sur le calendrier des évolutions que vous envisagez ?

le rôle des grossistes-répartiteurs est essentiel. Il importe qu'ils puissent continuer à assurer leur mission dans les meilleures conditions.

dont ils estiment qu'elle aurait pour effet d'assurer la pérennité du secteur de la répartition, viendrait en fait perturber l'équilibre économique global de la distribution des médicaments, sans présenter les garanties escomptées. La suppression d'une contribution qui assujettit aussi bien les laboratoires que les grossistes-répartiteurs ne serait pas de nature à favoriser davantage la répartition que la vente directe. Par ailleurs, nous avons calculé que cette mesure représenterait 75 millions d'euros de pertes de recettes pour l'assurance maladie. Nous y sommes donc défavorables. Nous nous sommes engagés à changer le modèle pour le premier trimestre

Il ne me paraît ni équitable ni opportun de prévoir un régime de taxation spécifique sur les vaccins, d'autant plus- le récent rapport du Sénat sur la pénurie de médicaments et de vaccins l'a montré -que les vaccins sont fréquemment touchés par des ruptures d'approvisionnement.

Cet amendement vise à favoriser la relocalisation en France de sites de production de médicaments et substances pharmaceutiques essentiels à la sécurité sanitaire de notre pays, conformément aux recommandations de la mission d'information du Sénat sur la pénurie de médicaments et de vaccins. vaccins. Il prévoit ainsi de mettre en place des abattements sur l'assiette des contributions prévues à l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, au bénéfice des entreprises pharmaceutiques s'engageant sur des investissements consacrés au développement de nouvelles capacités de production situées en France et destinées à produire des médicaments et substances pharmaceutiques actives considérées comme stratégiques pour les besoins de santé de notre population. Il est prévu que le dispositif soit limité dans le temps : les entreprises auront jusqu'au 31 décembre 2021 pour soumettre à l'administration fiscale leur plan d'investissement, afin de bénéficier de ces abattements pour une durée maximale de cinq ans. ? La question soulevée par les auteurs de cet amendement paraît en effet cruciale : la lutte contre les pénuries de médicaments doit certainement passer par une relocalisation des capacités de production de certains produits stratégiques. En l'état, la solution proposée ne paraît cependant pas nécessairement la plus incitative, et donc la plus efficace, en raison du faible montant de la contribution visée.